La séance est reprise. J'informe le Sénat qu'une candidature pour siéger au sein de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes a été publiée. Cette candidature sera ratifiée si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre règlement.

dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents. Je rappelle que l'auteur de la demande du débat dispose d'un temps de parole de huit minutes, puis le Gouvernement répond pour une durée équivalente.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, savez-vous, madame la secrétaire d'État, comment on remarque la bascule de la précarité à la pauvreté, puis à l'extrême pauvreté, chez nos concitoyens ?

Vous commencez par faire très attention à votre alimentation. Et « faire attention », ici, ce n'est pas manger des aliments de meilleure qualité. Au contraire, il s'agit d'acheter au moins cher : moins de viande, de plus en plus de pâtes, une alimentation de moins en moins variée avant d'aller chaque semaine au discount. Vous n'aviez déjà plus beaucoup de sorties culturelles. Musées et cinémas sont désormais bannis et votre seule sortie du week-end a lieu au centre commercial, non pas pour acheter, mais pour vous balader. Puis vient le jour où vous ne pouvez plus payer la cantine des enfants. Vous êtes donc obligé de les en retirer, alors que, pour beaucoup, c'était le seul repas équilibré de la journée. enfin le jour où, acculé dès le 15 du mois, vous êtes obligé de faire un choix cornélien : soit payer la facture d'électricité ou de gaz, soit payer le loyer. Vous faites le choix, qui n'en est pas un, de ne pas payer la facture d'électricité, car c'est souvent la moins importante et, surtout, vous pensez que vous pourrez la rattraper le mois suivant.

Vous ne savez plus vers qui vous tourner pour demander de l'aide. Telle est la situation de centaines de milliers de nos concitoyens chaque année. Je veux dire à celles et ceux qui sont dans ce cas qu'ils n'ont pas à avoir honte. Si le pouvoir politique a véritablement la main sur le pouvoir économique, c'est nous, ici même, qui devrions avoir honte. Comment se fait-il que, dans un pays qui est la sixième puissance mondiale, dans un pays où les grandes entreprises viennent de battre des records de versement de dividendes aux actionnaires- 57 milliards

En France, l'Observatoire national de la précarité énergétique dénombrait 12 millions de personnes en situation de précarité énergétique en 2016. Selon le médiateur de l'énergie, près de 30 % des Français admettent avoir restreint le chauffage pour alléger leur facture. Et le nombre de ménages qui se privent de chauffage est en constante augmentation, ce qui n'est pas sans conséquence sur la détérioration des logements et la santé. Selon l'Insee, les prix de l'énergie ont augmenté de 13,5 % entre l'été 2017 et la fin de 2018 et vont encore augmenter à l'été 2019. Or l'Observatoire national de la précarité énergétique rappelle qu'une augmentation de 10 % du prix de l'énergie ferait basculer 423 235 ménages supplémentaires en situation de précarité énergétique. Les inégalités de revenus se sont fortement creusées au cours de la dernière décennie et une hausse des prix de l'énergie est devenue insupportable pour beaucoup. Comment s'étonner, dans ce contexte, que des dizaines de milliers de nos concitoyens enfilent des gilets jaunes et occupent des ronds-points pour crier leur colère et exiger justice sociale et fiscale ? La question de la précarité énergétique est vaste : transition énergétique, fiscalité écologique, privatisation d'Engie, remise en cause des tarifs réglementés, augmentation de ces derniers, mobilité ... Il s'agit d'une problématique majeure qui va bien au-delà de sa définition légale, fondée sur la situation sociale et économique d'un ménage, sur l'état de son logement, sa qualité thermique et sa fourniture d'énergie. Certains facteurs de précarité sont clairement identifiés : augmentation du prix du pétrole et du gaz, libéralisation du marché de l'électricité, hausse des prix de l'immobilier et de la demande en énergie, stagnation des revenus, étalement urbain, remise en cause des services publics collectifs. La liste est loin d'être exhaustive. Nous ne pouvons en rester à ce constat. Si nous admettons que l'énergie est un bien commun de l'humanité, nous devons la sortir du secteur marchand. Je vais sûrement vous choquer,

ans que nous répondons avec servilité à ses injonctions de dérégulation, de mise en concurrence et de privatisation, les prix augmentent pour les usagers devenus des clients, les dividendes s'envolent- Engie est la deuxième

qui s'accélère avec votre gouvernement. Vous continuez, en liquidant les actifs de l'État dans Engie, en préparant le démantèlement d'EDF. En somme, en livrant le secteur de l'énergie, secteur d'intérêt général, au privé, dont l'objectif est la rémunération du capital, c'est-à-dire le profit, le profit, le profit ! Or comment répondre au défi de résorber la précarité énergétique et au défi d'avenir que représente la transition énergétique sans un secteur public répondant à un seul intérêt, celui de l'humain et de la planète ? Il faut des mesures fortes. La transition écologique passera aussi par une fiscalité écologique, qui a des effets sociaux les ménages ne sont pas touchés de la même façon. Souvent, ce sont les ménages les plus fragiles qui ont, proportionnellement à leurs revenus, les dépenses énergétiques les plus importantes. Taxer l'énergie revient alors à fragiliser davantage des populations déjà en difficulté. Lutter contre la précarité énergétique nécessite de mettre en place des politiques publiques ciblées sur les facteurs fragilisant les ménages : revenu disponible, prix de l'énergie et conditions de vie Cela passe par une remise en cause des politiques de libéralisation du secteur de l'énergie et des transports, qui ne s'est pas faite dans l'intérêt des consommateurs, mais seulement dans celui des actionnaires, et par un encadrement des prix de l'immobilier. Cela passe aussi par une intervention massive de l'État dans l'aménagement du territoire et la rénovation énergétique.

en droit fondamental. Les coupures d'énergie doivent être interdites tout au long de l'année pour les ménages en situation de précarité énergétique. Il n'est pas justifié, dans la France du XXI siècle, de couper l'électricité ou le gaz. De plus, la contribution au service public de l'électricité, ainsi que la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel, qui augmente progressivement chaque année, doivent être supprimées pour les ménages précaires.

augmenter les salaires, au lieu de pratiquer la charité à coup de chèques énergie, dont les gens ne veulent pas. Ils veulent une seule chose : être en capacité de payer eux-mêmes leurs factures. Il faut donc partager le gâteau de la richesse créée dans ce pays en augmentant les salaires

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Gay, ce débat est consacré à la précarité énergétique, devenue, vous avez malheureusement raison, une réalité pour nombre de nos concitoyens. La lutte contre la précarité énergétique est donc un enjeu important de nos politiques de transition énergétique et de lutte contre la pauvreté. Vous avez cité des données, je parlerai de celles de l'Observatoire national de la précarité énergétique : 11,9 % des Français ont consacré, en 2017, plus de 8 % de leurs revenus au chauffage, contre 13,8 % en 2013. Les progrès sont donc réels, mais extrêmement lents. L'enquête annuelle du médiateur de l'énergie montre que 15 % des répondants ont souffert du froid plus de vingt-quatre heures dans leur logement, 40 % d'entre eux en raison d'une mauvaise isolation. La précarité énergétique, ce sont des difficultés individuelles de ménages qui ne vivent pas bien, en tout cas pas dans un logement confortable, pour qui les dépenses de chauffage et de transports sont trop élevées et qui ont, vous l'avez rappelé, du mal à payer leur facture d'énergie. Pour répondre à cette situation d'urgence énergétique et sociale, le Gouvernement a déjà mis en place des aides dédiées et les améliore chaque année. En 2015, environ 158 000 ménages ont bénéficié d'une aide du Fonds de solidarité pour le logement pour payer leur facture d'énergie. On a dénombré, en 2017, près de 550 000 interventions des fournisseurs d'énergie à la suite d'impayés. Depuis 2017, nous avons renforcé ces mesures. Nous les renforcerons encore en 2019 et en 2020.

Indépendant du mode de chauffage, il est plus équitable que les anciens tarifs sociaux de l'électricité et du gaz, et les ménages le reçoivent automatiquement, dès qu'ils y sont éligibles. À l'automne 2018,

sur la rénovation. Notre objectif est de réaliser 500 000 rénovations énergétiques par an, dont 150 000 pour les passoires énergétiques du parc privé- les plus importantes -et 100 000 logements sociaux que nous rénovons avec le concours de la Caisse des dépôts et du grand plan d'investissement. Aujourd'hui, la France compte environ 7 à 8 millions de passoires énergétiques dont nous savons que la moitié est habitée par des ménages modestes ou très modestes. Plusieurs outils existent : le crédit d'impôt

année, l'ANAH a accompagné 62 000 rénovations dans le cadre de son programme Habiter mieux, soit près de 20 % de plus qu'en 2017. Son objectif est d'atteindre 75 000 rénovations aidées par an. Vous le savez, l'action de l'Agence permet de rechercher la synergie entre l'efficacité énergétique et d'autres axes d'intervention tels que la lutte contre l'habitat indigne ou le redressement de copropriétés en difficulté. Ces rénovations sont ambitieuses et ont un effet extrêmement positif en matière d'économies d'énergie : nous constatons en moyenne un gain de 40 %. Nous nous appuyons

L'obligation précarité énergétique dans le programme des C2E, entre 2018 et 2020, représente un investissement de près de 2 milliards d'euros sur trois

Nous travaillons aussi sur le financement complémentaire. En loi de finances pour 2019, nous avons très fortement simplifié l'éco-prêt à taux zéro, ou éco-PTZ, à la fois sur les types de travaux et sur les types de logements éligibles. Les C2E nous permettent également de mobiliser les banques pour faire en sorte qu'elles expliquent elles-mêmes à nos concitoyens les différentes aides dont ils bénéficient et la capacité à mobiliser des financements complémentaires. Nos efforts portent également sur le terrain de la mobilité. Vous avez cité l'étalement urbain, monsieur le sénateur, et il est vrai que, dans les territoires ruraux et périurbains, la voiture reste indispensable. Nous avons un double objectif de réduction des pollutions en termes de consommation de carburant et d'accompagnement des ménages les plus modestes. Je citerai uniquement la mise en place de la prime à la conversion pour les vieux véhicules 300 000 dossiers déposés en 2018, 255 000 traités et 71 % de ménages non imposables aidés à hauteur de 2 000 euros. Nous avons renforcé cette prime en 2019

En effet, ce crédit d'impôt, versé pour l'instant avec une année de décalage, constitue un facteur bloquant important pour les ménages modestes ou très modestes. Nous savons aussi que nous devons mieux informer les acteurs de la rénovation et les ménages.

Enfin, nous devons repenser l'organisation générale du service public de l'efficacité énergétique. Au regard du travail engagé avec Régions de France sur la définition précise de ses missions et sur ses modalités de financement, l'objectif est de proposer des solutions de mise en oeuvre nationale et des déclinaisons régionales à partir du troisième trimestre de 2019 dans des territoires pilotes. Nous devons venir à bout des passoires thermiques, en particulier dans le parc locatif privé. L'orientation retenue par la programmation pluriannuelle de l'énergie consiste à renforcer les aides pour les propriétaires bailleurs avant d'envisager d'éventuelles phases plus normatives. Dès lors, d'ici à 2021, la location d'un logement privé de catégorie F ou G ou la mutation d'un même logement seront soumises à la réalisation d'un audit énergétique. Pour accompagner cette obligation, il est d'ailleurs prévu de financer cet audit pour les ménages modestes, propriétaires de logements de type passoire énergétique. Nous savons que le chemin est long, que nous devons encore renforcer les moyens et imaginer d'autres formes d'intervention. Nous attendons aussi le retour des propositions issues du grand débat national en cours dont j'espère qu'elles amèneront de nouvelles idées concrètes. En tout cas, soyez assurés que la mobilisation de ce gouvernement pour la lutte contre la précarité énergétique est totale. Nous allons Je rappelle que chaque orateur dispose de deux minutes maximum pour présenter sa question, suivie d'une réponse du Gouvernement pour une durée équivalente. Dans le cas où l'auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de trente secondes supplémentaires, à

Les promesses n'engageant que ceux qui y croient, nous nous étions interrogés sur la portée réelle d'une telle annonce. Bien nous en a pris puisque, le 7 février dernier, la CRE a annoncé une hausse de 5,9 % des tarifs réglementés, au plus tard le 1 juin 2019. Malgré la réponse du ministre de Rugy à la question d'actualité que je lui avais posée le 14 février dernier, il s'agit bien d'une hausse payée par les ménages sur la facture d'électricité, au mois de juin ou à l'hiver prochains.

qui reproche à la CRE d'abuser de son pouvoir en faisant fi des lois existantes pour imposer par voie réglementaire ce qui relève du pouvoir législatif. Nous traversons donc une période puisque jamais deux autorités indépendantes, censées toutes les deux veiller et contrôler la concurrence, ne se sont trouvées publiquement en conflit. Face à cette cacophonie, le Gouvernement doit prendre position. Les Français doivent savoir où il se situe face à cette hausse annoncée des prix de l'énergie et en matière d'amélioration

secrétaire d'État. Madame la sénatrice, vous m'avez interrogée sur les tarifs réglementés de l'électricité. Je voudrais vous apporter quelques précisions. Comme vous le savez, les tarifs de l'électricité n'ont pas augmenté pendant l'hiver, comme le Gouvernement s'y était engagé à la suite à la crise que nous avons connue en octobre et novembre dernier. La prochaine augmentation sera donc appliquée, au plus tôt, le 1 juin. tôt, le 1 juin. Les formules sont fixées par la loi, en application des directives communautaires. Il n'existe aucun conflit entre les différentes autorités. L'Autorité de la concurrence n'a d'ailleurs pas dit que la CRE outrepassait son pouvoir sur le sujet. La parole

15 % des personnes interrogées ont déclaré avoir souffert du froid dans leur logement l'hiver dernier. En outre, un tiers des Français ont restreint leur consommation de chauffage, faute de revenus suffisants. Enfin, les ménages en précarité dépensent en moyenne 22 % de plus pour la facture énergétique de leur logement que la moyenne nationale. Nous connaissons donc les trois facteurs de la précarité énergétique : premièrement, la fragilité des foyers aux maigres ressources financières ; deuxièmement, la mauvaise isolation des logements ; troisièmement, le prix de l'énergie.

peut-être même la mise en place d'un fournisseur d'électricité universel de dernier recours et, enfin, le chèque énergie, renforcé et élargi à toutes les énergies. En ce qui concerne ce dernier, nous avions suggéré, par amendement, en décembre dernier, de faire plus- hélas, sans succès. Il faut donc renforcer les mesures curatives et préventives pour faire face à l'urgence, car si nous voulons agir efficacement sur le moyen et le long terme, il faut faire un immense effort en matière de rénovation thermique des logements.

le durcissement des obligations à la location des passoires thermiques, comme je l'ai indiqué dans mon intervention liminaire, nous commençons par mettre en place une obligation d'audit énergétique, ce qui permettra d'objectiver la situation de ces passoires thermiques avant leur mise en location, avant d'envisager des solutions plus normatives. Pour ce qui est du prix des énergies, comme je l'ai souligné, l'électricité n'a pas augmenté et le gaz a baissé au début de cette année. Enfin, nous avons étendu très fortement le chèque énergie, qui est passé de 3,6 millions à 5,8 millions de ménages éligibles

parole est à Mme Françoise Laborde. « Dès que le froid arrive, c'est le casse-tête qui recommence. On sait qu'il va falloir dormir tous dans la même pièce. J'ai acheté un radiateur à roulettes que je mets en route le soir quand les enfants rentrent de l'école. En journée, je me débrouille comme je peux, je vais dans des endroits chauffés, comme les galeries marchandes. Dans le salon il fait à peine 12 degrés, pour avoir chaud on dort ensemble ». Voilà l'extrait d'un témoignage du rapport de la Fondation Abbé Pierre, publié en février dernier. Face Face à ces situations de détresse, je tiens à souligner, avec l'ensemble de mes collègues du groupe du RDSE, le rôle central des collectivités territoriales pour soutenir, sur le terrain, les ménages en difficulté : les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, les conseils départementaux, les régions et les métropoles sont des tiers de confiance, en première ligne, impliqués dans la conduite de politiques de prévention avec, par exemple, la construction ou la rénovation du parc de logements sociaux à basse consommation énergétique.

au logement. Un impayé d'énergie est un facteur aggravant pour les ménages les plus fragiles. Commence alors le cercle vicieux des arbitrages impossibles de la vie quotidienne tels que choisir entre manger ou se chauffer. Il faut dire que la part du logement dans le budget des ménages est passée de 9,3 % en 1959 à plus de 22 % aujourd'hui. En outre, 60 % des ménages les plus pauvres sont contraints par les dépenses fixes, contre 35 % pour les classes moyennes et aisées. La vulnérabilité énergétique des classes populaires est désormais posée dans l'agenda social. Sans préfigurer les conclusions du grand débat national, quelles mesures compte prendre le Gouvernement pour alléger la charge financière des millions de ménages les plus précaires énergétiquement

la contractualisation entre l'ANAH et les collectivités territoriales. L'Agence contractualise aujourd'hui avec environ 70 % des collectivités territoriales- communes ou intercommunalités -pour accompagner ces politiques, les démultiplier

je souhaite attirer votre attention sur la forte augmentation, ces dernières années, des tarifs de l'abonnement « effacement jour de pointe », ou EJP, proposé par EDF. Cet abonnement, je le rappelle, permet aux consommateurs de bénéficier d'un tarif d'électricité avantageux la majorité de l'année, hormis certains jours en automne et en hiver, où ce tarif augmente fortement. Cet abonnement est profitable tant aux consommateurs, qui allègent leur facture, qu'au fournisseur d'électricité, qui profite de leur consommation réduite au cours des 22 « jours de pointe L'abonnement « effacement jour de pointe » n'est plus disponible à la vente depuis 1998, et seules les personnes l'ayant souscrit antérieurement à cette date ont encore le droit d'en bénéficier. Toutefois, pas moins de 450 000 foyers l'utilisent encore, et c'est d'ailleurs par des abonnés que j'ai été alerté d'une augmentation des tarifs. En effet, on assiste depuis plusieurs années à une augmentation continue de l'option EJP pour les « jours classiques a été de 6,5 %. Parallèlement, on constate une baisse du prix des tarifs les « jours de pointe ». Le tarif de l'électricité pour les « jours classiques » ayant quasiment rejoint celui d'autres abonnements, l'option EJP est de plus en plus dénuée d'intérêt. Plusieurs arguments plaident en faveur de la préservation d'un tarif EJP distinct du tarif de base. Premièrement, il est à craindre qu'une telle augmentation mette certains abonnés en situation de précarité énergétique. Deuxièmement, le tarif EJP permet de baisser la demande d'énergie pendant les « jours de pointe », où la consommation est la plus forte et où l'offre peine parfois à suivre la demande. Enfin, troisièmement, ce système s'inscrit pleinement dans les engagements pris par notre pays en matière de réduction de sa consommation d'énergie. Par conséquent, ne pensez-vous pas, madame la secrétaire d'État, qu'il serait pertinent de ne pas priver d'effet l'option EJP, à moins d'offrir une alternative aux abonnés ?

L'option EJP, ou « effacement des jours de pointe », a été mise en place en 1982. Il s'agit d'un tarif à effacement destiné à faire baisser la consommation lors des jours de pointe, soit vingt-deux jours par an, avec dix-huit heures de pointe dans chacune de ces journées, choisies la veille pour le lendemain en fonction des prévisions de court terme de la demande et de la disponibilité des moyens de production. Pendant ces jours de pointe, le prix de l'électricité est plus cher, pour inciter à une diminution, voire à un effacement, de la consommation. Les autres jours, le prix de l'électricité est plus faible que la moyenne. La création de l'option Tempo en 1996 poursuivait la même logique que l'option EJP, en offrant des prix contrastés selon un découpage en trois types de jours. Cette option a permis une avancée dans le domaine de la flexibilité, en permettant une gestion plus fine des incitations, mieux à même de s'adapter aux variations de prix sur toute l'année, alors qu'EJP propose une approche plus simple, sur vingt-deux jours de pointe. En 1997, EDF et l'État ont considéré qu'il n'était pas nécessaire de faire coexister ces deux offres à effacement dans l'option des tarifs réglementés de vente, et l'option EJP, comme vous l'avez signalé, a été mise en extinction. Aucune nouvelle souscription n'est donc plus possible depuis 1997. Il faut savoir que ces deux options, EJP comme Tempo, ne sont pas des outils de lutte contre la précarité énergétique. Ce sont des outils permettant de limiter la consommation les jours de grande tension sur le système électrique. Ils peuvent néanmoins permettre aux ménages de réduire leur facture, si ces derniers sont prêts à faire des efforts significatifs de flexibilité sur leur consommation. Ces efforts sont facilités par le développement des équipements connectés et pilotables à distance. Vous m'alertez sur l'évolution des tarifs EJP, à laquelle je porterai une attention particulière. En attendant, le ministère conduit des études avec l'Ademe et la CRE, pour voir s'il y a un intérêt à développer davantage ces types d'effacement dits tarifaires et définir les outils à développer pour ce faire. La parole

La pauvreté et l'accès à un logement décent font partie depuis longtemps des politiques publiques, mais la question de l'énergie est plus récente et trouve sa définition officielle dans la loi Grenelle II de 2010. Cette précarité est un facteur aggravant de la pauvreté, qui va bien au-delà du mal-logement. Elle pousse les ménages au surendettement, sans compter que le manque de chauffage est également dangereux pour la santé physique et psychologique. Certes, des dispositifs existent pour limiter cette précarité et des fonds européens dédiés aux collectivités locales permettent de financer l'isolation des appartements HLM anciens, mais également des propriétés dégradées. Pour exemple, la communauté d'agglomération Melun Val de Seine a permis à l'office public départemental de recevoir un million d'euros, soit 50 % du coût de la rénovation thermique de 234 logements. Cela devrait représenter 30 % d'économies sur les charges de chauffage des locataires. La précarité énergétique est l'un des sujets sur lesquels l'écologie s'accorde le mieux avec l'économie. Parvenir à mieux utiliser l'énergie, pour en consommer moins, voilà qui serait bon pour le pouvoir d'achat et l'environnement. Madame la secrétaire d'État, m'appuyant sur une recommandation formulée le 29 janvier dernier dans un rapport d'information parlementaire,

et, plus généralement, au mal-logement. Vous avez raison, cette notion a été définie dans la loi Grenelle II. C'est important, parce que cela permet de nommer la difficulté et, donc, de la traiter. Vous avez évoqué les situations de surendettement. C'est la raison pour laquelle nous insistons aujourd'hui sur le travail avec les banques, à la fois pour qu'elles soient en état de repérer ces situations, mais aussi de proposer des solutions à leurs clients, solutions financées par la puissance publique au travers du CITE ou des programmes d'économie d'énergie, et et cofinancées par elles-mêmes au travers d'un prêt à taux zéro amélioré. L'exemple de Melun Val de Seine montre qu'il est effectivement possible de concilier écologie et économie. La politique de rénovation bénéficie

Ce sont des jeunes, des retraités, des inactifs, qui vivent dans de véritables passoires thermiques et consacrent plus de 10 % de leurs revenus aux dépenses d'énergie.

? J'aimerais également vous alerter sur le fait que certains bailleurs n'investissent pas dans la rénovation énergétique de leur bien, profitant de la pauvreté de leurs locataires. Comment remédier à une telle

qui sera, l'année prochaine, transformé en prime pour les ménages les plus modestes et fusionné avec les aides de l'ANAH. La question posée est bien celle de la lisibilité, de la transparence et de la garantie données à toutes ces aides. C'est la raison pour laquelle nous massifions les programmes de rénovation financés par les certificats d'économie d'énergie, désormais portés par les grands énergéticiens eux-mêmes, qui sont en mesure de convaincre leurs clients du sérieux et de la réalité de ces aides. C'est également la raison pour laquelle nous développons le programme Faire, qui est une plateforme destinée à tous les acteurs. Il doit permettre de créer un label reconnu par nos concitoyens et par les professionnels, pour porter des offres garanties par l'État et de qualité. C'est enfin la raison pour laquelle nous travaillons, depuis la loi de 2015, en reprenant cette réflexion avec Régions de France, sur la mise en place d'un service public de l'efficacité énergétique, qui nécessite la simplification des guichets, voire le passage à un guichet unique, mais aussi la capacité à certifier l'existence de tiers de confiance, qui sont seuls capables de convaincre nos concitoyens de mener des actions de rénovation. La parole

bien évidemment, madame la secrétaire d'État, dans le prolongement des questions qui viennent de vous être posées. La précarité énergétique s'est imposée, en France, comme un sujet de préoccupation majeur. Selon l'Observatoire national de la précarité énergétique, 6,7 millions de Françaises et Français dépensent plus de 8 % de leurs revenus dans l'énergie. Au cours de l'hiver dernier, 15 % des ménages ont affirmé avoir souffert du froid dans leur domicile. Les raisons évoquées ? Des défauts d'isolation dans 40 % des cas et/ou un manque de chauffage. Un ménage sur quatre est en situation de vulnérabilité énergétique, avec une surreprésentation des ruraux, des agriculteurs et des retraités. Afin de limiter les effets de la précarité énergétique, un certain nombre de dispositifs ont été mis en place par le législateur. Les tarifs sociaux de l'énergie ont été remplacés en 2018 par un chèque énergie d'un montant moyen de 150 euros. Il a été perçu par 3,6 millions de ménages.

être alloués. Mais tous n'y ont pas recours, parfois par manque d'information. Ma question est donc la suivante : quels sont les moyens développés aujourd'hui afin de mieux informer les ménages en situation de précarité énergétique sur tous ces dispositifs ?

Les questions du non-recours et de l'information sont donc extrêmement importantes dans cette politique, à la fois de lutte contre la précarité énergétique par le soutien du pouvoir d'achat, mais aussi de rénovation.

Toutefois, 93 % des bénéficiaires affirment qu'ils ont compris le dispositif et qu'ils savent s'en servir. Au-delà du chèque énergie, il y a l'accès au programme

plus loin, en sensibilisant les ménages modestes au fait qu'ils peuvent avoir accès à ce programme. Tel est l'objectif de la plateforme FAIRE, que je citais dans mon propos précédent. Enfin, nous mettons une partie de l'argent des certificats d'économie d'énergie dans des programmes d'accompagnement. Je vous ai cité celui qui concerne les banques,

Ce programme d'information permet de sensibiliser les ménages en situation de précarité énergétique, pour qu'ils puissent avoir accès à la rénovation. La Poste mène également un travail de proximité, pour permettre à tous ses clients de

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la veille du dépôt du projet de loi Énergie, le Gouvernement a décidé de revoir sa copie, jugeant le texte trop peu ambitieux sur le climat. Ce report intervient alors qu'est déposé aujourd'hui un recours au tribunal administratif pour inaction climatique, dans un contexte de mobilisation citoyenne sans précédent en faveur du climat, lancée par la jeune Suédoise Greta Thunberg. L'avis du Conseil national de la transition écologique, le CNTE, dont j'ai l'honneur d'être membre, était pour le moins réservé sur ce projet de loi qui entérine des reculs importants par rapport à la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. En effet, le texte n'aborde pas la question centrale qui nous réunit ici, à savoir la lutte contre la précarité énergétique, laquelle est au coeur du nouveau contrat social et écologique à mettre en place. Madame la secrétaire d'État, les deux questions sont intimement liées. Nous sommes heureux de constater que le Gouvernement, après avoir développé pléthore d'éléments de langage, considère maintenant qu'il lui faut revoir sa copie. J'espère que cette révision vous permettra, madame la secrétaire d'État, de prendre en compte les remarques du CNTE, qui vous invitait à « instaurer le service public de performance énergétique de l'habitat

L'Autorité environnementale vient de rendre un avis acerbe sur le manque d'ambition du Gouvernement s'agissant du plan de rénovation thermique. Selon cette instance, 15 milliards à 30 milliards d'euros devraient être dépensés chaque année pendant trente ans pour rattraper le retard pris. Au-delà du manque de financement, l'absence de structuration du service public de performance énergétique fait courir un très grand risque aux ménages, qui peuvent être confrontés à des maîtres d'ouvrage indélicats, que les associations de consommateurs ne cessent de dénoncer.

la neutralité carbone en 2050. C'est plus que l'objectif précédent, à savoir une division par quatre de nos émissions de gaz à effet de serre. Je sais que ce sujet a pu donner lieu à certaines incompréhensions. C'est la raison pour laquelle nous allons clarifier ce point. La neutralité carbone en 2050 suppose une réduction de nos émissions par

entre les régions, les départements, les communes, les intercommunalités et l'État. Tel est l'objet du travail qui commence dans trois régions pilotes. Il doit nous permettre de trouver la meilleure organisation possible au service de nos concitoyens. La parole

contexte de vulnérabilité financière des ménages aux plus faibles revenus, l'indicateur du « taux d'effort énergétique » par rapport aux revenus

très concrètement, que comptez-vous faire, madame la secrétaire d'État, pour combler les failles du dispositif s'agissant de la non-utilisation par les bénéficiaires des attestations leur permettant d'avoir recours à des droits protecteurs

? La parole est à Mme la secrétaire d'État. Madame la sénatrice, vous m'avez interrogée sur la manière dont on peut accompagner les ménages les plus vulnérables. Il s'agit effectivement de l'un de nos objectifs de politique publique en matière de lutte contre la précarité énergétique. C'est bien la raison pour laquelle nous avons mis en place le chèque énergie, qui remplace les tarifs sociaux de l'électricité et du gaz, ce chèque énergie étant à la fois plus juste et plus simple d'utilisation. D'abord, les ménages éligibles le sont sur la base de leurs revenus, donc indépendamment de la réalité de leur effort, pour tenir compte du fait que, comme vous le signalez, certains ont simplement abandonné leur capacité à se chauffer et donc à consommer. Mais ce sont bien tous les ménages modestes qui sont accompagnés. Nous avons augmenté le seuil de revenus pour l'éligibilité à ce chèque énergie, ce qui nous permet de viser

nous n'avons pas revu nos ambitions à la baisse dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie, pas plus que dans la loi Énergie qui vient d'être citée, puisque nous maintenons notre ambition de 500 000 rénovations par an. Nous maintenons

Cette disposition permettait d'accorder une déduction forfaitaire pouvant aller jusqu'à 140 euros par an, selon la puissance souscrite et la composition familiale. Ce dispositif était entièrement automatisé. Les charges induites par la mise en oeuvre du dispositif TPN pour les fournisseurs d'énergie faisaient l'objet d'une déclaration au régulateur, la CRE, et étaient financièrement compensées. Des champs spécifiques étaient prévus dans la déclaration à cet effet. Depuis janvier 2018, un nouveau dispositif appelé chèque énergie, institué par décret du 6 mai 2016, a été mis en place et s'est substitué au TPN après deux années d'expérimentation. Il s'agit d'un moyen de paiement qui est distribué aux bénéficiaires par l'Agence de services et de paiement, l'ASP, suivant un calendrier prédéfini par la région. Ce dispositif n'est pour l'instant pas entièrement automatisé, car les bénéficiaires adressent leur chèque énergie au format papier, ce qui entraîne pour les fournisseurs des charges de gestion administrative et de traitement des appels téléphoniques. Pour ce nouveau dispositif, aucune rubrique n'est prévue dans le formulaire de déclaration de la CSPE au régulateur, pour se faire compenser ces charges supplémentaires. Madame la secrétaire d'État, comment comptez-vous remédier à cette situation, qui nécessite une compensation des charges induites ? Ces dernières seront amplifiées en 2019 par l'augmentation du nombre de bénéficiaires du chèque énergie, qui devrait passer de 3,6 millions à 5,8 millions au niveau national ? La parole est à Mme la secrétaire

Néanmoins, il est perfectible, vous avez raison, les uns et les autres, de le rappeler. Nous travaillons dans trois directions pour l'amélioration de ce dispositif, certaines actions ayant déjà été mises en place. D'abord, il s'agit de la possibilité d'utiliser le chèque énergie pour payer en ligne. Le chèque devient donc un moyen de paiement pour 30 % de ses utilisations, pour les fournisseurs qui ont déjà réalisé les développements nécessaires. nous organisons également la possibilité de préaffecter le chèque directement au fournisseur. Environ 600 000 demandes ont eu lieu au titre de la campagne de 2018. Dans ce cas, le bénéficiaire reçoit non plus directement son chèque, mais simplement un courrier lui rappelant son choix de préaffectation, accompagné des attestations nécessaires. Enfin, nous prévoyons la possibilité, à compter de la campagne de 2019, de préaffecter également l'attestation,

Les flux sont signés pour les fournisseurs les plus importants et la remise dématérialisée sera disponible dans les prochaines semaines pour les plus petits. Nous sommes donc attentifs à faire évoluer le dispositif, pour répondre au mieux aux attentes et aux enjeux des personnes les plus démunies, pour un coût le plus juste possible. La parole est à Mme Angèle

calfeutre son habitat, on vit dans une pièce unique ou on s'endette pour payer son électricité, c'est devenu une réalité dans notre pays. Aujourd'hui, le fait d'être locataire est de plus en plus un indice de situation financière délicate. Parmi les ménages concernés, certains n'accéderont jamais à la propriété ; ils sont et seront toujours captifs d'un marché insuffisamment réglementé. Ce débat est donc l'occasion de se pencher sur le cas particulier des locataires en situation de précarité énergétique. Les difficultés financières conduisent ces personnes à se tourner vers les loyers les moins onéreux, les moins-disants du marché, c'est-à-dire vers les habitats qui ont une mauvaise performance énergétique, ceux qui correspondent souvent aux classes F et G du diagnostic de performance énergétique, le DPE. Mal isolées, humides, voire dégradées, ces résidences font exploser la part du budget de ces ménages consacrée aux factures énergétiques. vous n'êtes pas sans le savoir, en ce moment même, des familles ne se chauffent pas et renoncent à l'eau chaude. Certes, le système actuel apporte des réponses- chèque énergie, aides sociales,

peuvent rester sourds aux demandes des locataires, qui n'ont ni le choix de changer d'habitat ni les moyens légaux de contraindre leur bailleur à engager les travaux nécessaires. Eh oui ! Face à ce défi majeur pour notre société, en proie à une crise profonde et dans laquelle la justice sociale est plus que jamais au coeur du débat,

ne pas avoir préconisé le plafonnement des loyers des habitations classées F ou G, sur un modèle similaire à celui de l'encadrement des loyers ? Nous sommes dans une triple problématique d'urgence sociale, climatique et énergétique ; nous serons très attentifs à la future loi relative à l'énergie.

cours du grand débat national, leur attachement à la transition énergétique, pour eux-mêmes, pour leurs enfants et pour la survie de notre planète. Il n'en demeure pas moins que les travaux liés au logement ont un coût substantiel, et que les prêts consentis pour financer, par exemple, des travaux d'économie d'énergie restent des prêts à rembourser, fussent-ils à taux zéro,

! , la bonne volonté des ménages, conjuguée aux facilités octroyées par le Gouvernement, se trouve réduite à néant, faute d'avoir un reste à vivre digne et de pouvoir emprunter, même à taux ma question : pour optimiser encore le système en faveur des ménages les plus précaires, l'État pourrait-il se substituer au débiteur pour ce qui concerne son assurance de prêt et la garantie demandée par les organismes de crédits ? La parole

C'est la raison pour laquelle le premier objectif de nos politiques publiques est de réduire le reste à charge, en particulier pour les ménages modestes. D'où deux mesures, dont je parlais. La première consiste en la concentration des certificats d'économies d'énergie, afin d'avoir des offres à un euro- chaudière à un euro,

Dans ses recommandations, cette organisation enjoignait aux États membres de l'Union européenne d'agir en faveur de l'allégement de la précarité énergétique dans les transports. Cette vulnérabilité énergétique est donc une réalité, à l'heure où 40 % des dépenses énergétiques des Français sont consacrées à l'achat de carburant. Dans la région Occitanie, l'une des plus vastes de France, la politique ferroviaire doit être un levier pour lutter contre la vulnérabilité liée à la mobilité. Le maintien des petites lignes et l'investissement dans les transports en commun du quotidien

À titre d'exemple, il serait intéressant d'ouvrir la gestion de certaines lignes du réseau ferré national aux collectivités locales ou de permettre aux communes et à leurs groupements de mettre en place une tarification de stationnement spécifique pour les personnes en situation de vulnérabilité économique, sur le modèle des tarifications solidaires pouvant être prévues pour l'usage des transports publics.

nous renforçons notre action selon plusieurs axes. Le premier consiste à penser une mobilité plus durable et accessible à tous. Pour ce faire, nous avons tenu les assises de la mobilité, auxquelles les collectivités ont été très largement associées, sous l'égide de Mme Élisabeth Borne, dont le projet de loi d'orientation des mobilités sera bientôt discuté au Sénat. Ce projet Ce projet de loi pose le principe de la généralisation des autorités organisatrices de la mobilité sur tous les territoires, pour développer de façon homogène les offres de mobilité, et il prévoit des mesures favorisant des mobilités actives, telles que le vélo, le covoiturage ou les véhicules en autopartage. Dans le cadre du grand débat,

Nous avons aussi beaucoup travaillé pour renforcer les actions concrètes et soutenir les personnes dans leur choix de mobilité. Je veux à cet égard redire un mot de la prime à la conversion, dispositif qui a été sensiblement renforcé en 2018, notamment au travers des véhicules éligibles et du montant des primes. Ce dispositif a connu un grand succès, avec près de 300 000 demandes et 255 000 dossiers déposés en 2018. En outre, 71 % des bénéficiaires sont non imposables, ce qui montre bien que la cible de nos concitoyens les plus modestes est atteinte. Nous allons encore renforcer ce dispositif en 2019,

est encore un peu trop tôt pour avoir un bilan de ce dispositif, cette « super-prime à la conversion », mais son démarrage est extrêmement encourageant. Enfin, nous mobilisons là encore les programmes de C2E, pour accompagner les ménages

et ainsi contribuer aux objectifs fixés par le Gouvernement en ce domaine. Si ce dispositif est vertueux dans son modèle, il reste en pratique vicié et, par conséquent, peu efficace.

Or, pour gagner en efficacité et éviter tout refus, ne faudrait-il pas que le fournisseur se charge lui-même du contrôle de l'éligibilité du consommateur ? En outre, du fait d'une information peu claire, les ménages peuvent difficilement faire jouer la concurrence ; on a d'ailleurs pu constater sur le territoire dont je suis élu jusqu'à 900 euros d'écart pour une même opération. De plus, le montant de la prime est calculé sur la base d'un gain moyen d'énergie, estimé par l'administration, et non sur le gain réellement obtenu grâce à une action d'économie d'énergie.

étant payés par les vendeurs d'énergie qui les rachètent, ces coûts sont répercutés sur les factures d'énergie des consommateurs. Comme trop souvent avec les aides à la rénovation énergétique, les locataires sont les grands perdants, car ils sont contributeurs, mais non bénéficiaires. Aussi, ne faudrait-il pas plutôt inciter les bailleurs aux travaux, un système de bonus-malus ? Enfin, après dix ans, le C2E reste un dispositif encore peu connu et donc peu utilisé, les pouvoirs publics faisant davantage la promotion des aides publiques- TVA à taux réduit ou CITE -, alors même qu'ils sont cumulables. Veuillez conclure. Vous arguez sans cesse de la nécessité d'une rénovation énergétique efficace, mais les moyens offerts restent peu lisibles et trop contraignants à mettre en place. Comment comptez-vous pallier cette difficulté ?

40 000 interventions sur les murs ou le plancher, 46 000 interventions sur des chaudières collectives, 43 000 changements de chaudière à condensation et 250 000 fenêtres. Il s'agit donc d'un dispositif massif, vous avez raison de le souligner, et il est financé de façon extensive.

La précarité énergétique des ménages nous touche au quotidien, surtout lorsque nous sommes maires et en contact avec les ménages en détresse. Nous devons faciliter la rénovation

mais, malgré une dizaine de tentatives, le site ne reconnaît pas mon numéro fiscal. Je contacte alors l'assistance par courriel ; j'attends encore que l'on me rappelle. Je contacte alors le numéro vert, qui me dirige vers le service de l'Orne ; j'ai beaucoup de chance, celui-ci tient une permanence une fois par semaine, le jeudi jusqu'à midi et il

de continuer d'améliorer l'accès à l'information. L'accès au système peut d'ailleurs également passer, pour les certificats d'économie d'énergie, par le biais des grands fournisseurs d'électricité ou de gaz.

l'augmentation du prix de l'essence s'inscrit dans la précarité énergétique. Nous pensons notamment à nos concitoyens qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture pour aller au travail, à ceux qui sont en zone blanche des transports publics-

il faut d'urgence augmenter les salaires dans ce pays, à commencer par le SMIC, en ouvrant des négociations dans chaque branche salariale pour tirer les rémunérations vers le haut, afin que les gens puissent vivre dignement et payer leurs factures.

tout un objectif de profit ? Nous ne sortirons pas les gens de la précarité énergétique si tous les secteurs de l'énergie sont libéralisés, ouverts à la concurrence, privatisés. En quatrième lieu-

Cette proposition de résolution, largement cosignée par plus de cent sénateurs et sénatrices, de groupes divers, illustre la participation du Sénat à une mobilisation dans laquelle se sont déjà inscrits le Parlement européen et l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. L'inscription de cette proposition de résolution à l'ordre du jour de notre assemblée est un acte fort qui fait écho à la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars, à la Journée onusienne de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines, célébrée le 6 février, et à la Journée internationale de la fille, inscrite à l'agenda de l'ONU depuis 2012. L'actualité récente conforte notre délégation dans ses choix

; le lancement, par la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, dix jours précisément avant cette séance, d'un plan pour éradiquer l'excision. Nous ne pouvons que nous réjouir, monsieur le secrétaire d'État, de cette convergence entre le Sénat et le Gouvernement dans la lutte contre ce scandale qui fait chaque année, dans le monde, trois millions de victimes : des femmes, des jeunes filles et des fillettes, parfois même des nourrissons de quelques jours. Toute leur vie, ces femmes seront durement affectées par ces pratiques barbares. Monsieur le secrétaire d'État, la délégation aux droits des femmes du Sénat, par ma voix, vous rappelle sa disponibilité pour travailler ensemble sur nos conclusions. Ce fléau sévit bel et bien sur notre territoire. Il menace des adolescentes qui fréquentent nos établissements scolaires et qui risquent, à l'occasion de congés passés dans le pays d'origine de leur famille, de se retrouver excisées, puis mariées contre leur gré. On sait par ailleurs que des mineures excisées accouchent dans nos hôpitaux. Quelques chiffres effrayants : toutes les sept secondes dans le monde, une fille de moins de 15 ans est mariée contre son gré le mariage forcé concerne, chaque année, 12 millions de filles de moins de 18 ans. À un âge où elles devraient aller à l'école et jouer, ces filles sont confrontées à l'horreur du viol conjugal et à des grossesses auxquelles leur organisme n'est pas adapté. Une fille sur cinq donne naissance à son premier enfant avant 18 ans. Les grossesses et les accouchements précoces causent chaque année 70 000 décès dans le monde. Les complications de la grossesse et de l'accouchement sont la deuxième cause de décès des filles de 15 ans à 19 ans. Les effets de ces grossesses précoces sont effroyables sur la santé des enfants. Hélas, le fléau du mariage des enfants n'est pas en voie de régression, bien au contraire. La multiplication des zones de crises humanitaires conduit certains parents confrontés à la misère et à l'endettement à souhaiter marier leurs filles, même très jeunes. Le mariage des enfants aggrave la pauvreté. La mobilisation contre le mariage des enfants dans le cadre de la présidence française du G7, qui a inscrit à son ordre du jour la question de l'éducation des filles, doit être généralisée. Je souhaite saluer, cet après-midi, l'engagement de celles et ceux- professionnels et bénévoles, hommes et femmes -qui oeuvrent chaque jour pour lutter contre des pratiques inacceptables que le relativisme culturel ne saurait justifier. Notre délégation plaide régulièrement pour que les structures engagées contre les violences faites aux femmes, et principalement les associations, disposent de moyens en cohérence avec l'ampleur des besoins. J'espère, monsieur le secrétaire d'État, que nous serons enfin entendus Pour conclure, je remercie nos collègues sénateurs qui ont signé cette proposition de résolution. Les combats que mène la délégation aux droits des femmes, nous en sommes convaincus, ne rencontreront le succès que s'ils sont aussi portés par des hommes. ! Le fait que quarante sénateurs aient rejoint notre initiative est un signal encourageant. La lutte contre les violences est un enjeu de société et non une affaire de femmes. Merci à vous, chers collègues ! Il me reste donc à vous demander de faire en sorte, par votre vote, que cette proposition de résolution devienne une résolution du Sénat. Certes, ce vote ne suffira pas à éradiquer les fléaux contre lesquels nous nous élevons, mais ce serait un signal fort donné par notre institution à ces victimes innombrables et à toutes celles et ceux qui s'engagent partout dans le monde pour les défendre et les accompagner. La parole

quelques jours après la Journée internationale des droits des femmes. Ce texte représente l'aboutissement de plusieurs travaux de la délégation aux droits des femmes, dont un rapport sur les mutilations sexuelles féminines dont j'ai eu le plaisir d'être corapporteure avec ma collègue Maryvonne Blondin. Annick Billon a rappelé les statistiques effroyables associées au mariage des enfants et aux grossesses précoces. Pour sa part, l'excision fait une victime toutes les quinze secondes dans le monde. En ce qui me concerne, je souhaiterais présenter les principales conclusions du rapport de la délégation aux droits des femmes sur les mutilations sexuelles féminines. Le rapport de la délégation se fonde sur des rencontres avec des victimes de mutilations, ainsi qu'avec des acteurs de la lutte contre l'excision. Permettez à l'élue des Yvelines que je suis de saluer le travail accompli par Women Safe, ex-Institut en santé génésique de Saint-Germain-en-Laye, pour accueillir et soigner les victimes. Très bien ! Les responsables de cet établissement exceptionnel nous ont accompagnés pendant nos travaux, comme d'ailleurs de nombreux autres acteurs. À travers les témoignages bouleversants des victimes avec lesquelles nous avons pu échanger, nous avons compris que l'excision n'est bien souvent qu'une des terribles épreuves jalonnant un long parcours de violences marqué par les mariages précoces ou forcés. À titre d'exemple, parmi les jeunes femmes accueillies au foyer « Une femme, un toit » dédié à l'hébergement de jeunes femmes victimes de violences, 80 % de celles qui ont subi une excision ont été mariées de force ou menacées de mariage forcé. Comme l'a dit notre présidente, nous avons noté l'annonce par le Gouvernement d'un plan d'ici à l'été pour éradiquer l'excision, ce qui va dans le sens de notre proposition de résolution. Nous serions donc heureux que celui-ci puisse s'inspirer de nos travaux, s'appuyer sur nos propositions et recommandations, ... Tout à fait ! ... car il faut aller au-delà des campagnes de communication sur les réseaux sociaux pour avancer sur ces sujets, monsieur L'une de nos recommandations vise ainsi à envisager un recensement systématique, dans les établissements d'enseignement secondaire, des jeunes filles qui quittent le collège à l'âge de l'obligation scolaire sans que l'établissement ait édité une autorisation de sortie ou. En effet, les jeunes filles concernées peuvent être de potentielles victimes d'excision ou de mariage précoce ou forcé dans le pays d'origine de leur famille. Une autre recommandation concerne les personnels de l'éducation nationale. L'enjeu de leur formation, qui nous paraît incontournable, est notamment de protéger les jeunes filles menacées d'excision ou de mariage forcé à l'occasion des congés scolaires. Dans le même esprit, notre rapport rappelle l'urgence d'un renforcement des moyens de la médecine scolaire, indispensable au repérage des victimes et à la protection des petites filles et adolescentes menacées d'excision. À bien des égards, les professionnels de santé appartenant à la communauté éducative- médecins, infirmières, psychologues -sont en première ligne pour contribuer au repérage et à l'orientation des victimes potentielles, qu'il s'agisse de l'excision ou du mariage forcé. Une autre recommandation invite à un signalement des mineures excisées qui accouchent en France, car ces jeunes filles ont pu être victimes de mariage forcé.

Dans ma pratique, j'ai été conduite à soigner de très jeunes filles, enceintes et mutilées : il n'y a pas d'histoire d'amour dans ce contexte, je vous le garantis ! On y trouve en revanche la litanie du mariage forcé et du viol conjugal, sans oublier les mutilations. » Dans ce Dans ce contexte, nous sommes fiers que, sur l'initiative de plusieurs membres de la délégation, l'une des recommandations de notre rapport ait trouvé une traduction législative dans la loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes pour étendre les missions de l'aide sociale à l'enfance au « repérage et à l'orientation des mineurs victimes ou menacés de violences sexuelles, notamment des mineures victimes de mutilations sexuelles Plus généralement, nous soulignons l'importance de la convention d'Istanbul, qui engage explicitement les États à sanctionner les mutilations et les mariages forcés. Le rapport appelle donc à une très large ratification de cet instrument international indispensable à la lutte contre toutes les violences faites aux femmes. Ma collègue Maryvonne Blondin vous en parlera tout à l'heure. Nous proposons aussi de marquer notre soutien aux associations qui agissent au quotidien contre les mutilations sexuelles féminines, dans un contexte financier trop souvent difficile. Nous souhaitons que ces subventions soient davantage prévisibles, dans une logique pluriannuelle. Nous appelons donc au renforcement des moyens alloués aux associations qui oeuvrent contre les violences faites aux femmes, sans nous limiter aux fléaux qui nous réunissent aujourd'hui. Je veux ici leur rendre hommage pour leur action décisive et saluer leurs représentants présents aujourd'hui dans les tribunes. Mes chers collègues, je vous remercie de votre attention et vous invite à voter cette proposition de résolution sans aucune hésitation. La parole

la rédaction de ce projet de résolution à partir du rapport que Marta de Cidrac et moi-même avons réalisé en mai 2018. Je salue aussi le travail de celles et ceux qui accompagnent

sobres et pudiques, mais ô combien chargées de souffrances, nous disant le choc terrible ou le néant complet après le « charcutage » qu'elles ont subi et leur reconnaissance envers tous ceux qui les ont aidées.

Si trente pays sont particulièrement concernés à l'instar de l'Égypte ou de la Somalie, l'excision ne constitue pas une problématique purement étrangère

contre les trois phénomènes distincts, mais bel et bien liés entre eux : les mariages des enfants, les grossesses précoces et les mutilations sexuelles féminines. Ils sont liés, car ils s'inscrivent dans un parcours véritable de l'ensemble des violences faites aux filles et aux femmes. Véritable violation des droits humains fondamentaux, du droit à l'intégrité physique et mentale, à la santé, les mutilations sexuelles féminines constituent l'expression même de la domination masculine sur le corps des femmes et leur sexualité. D'ailleurs, la délégation aux droits des femmes a préféré, à juste raison, l'expression « mutilations sexuelles à celle de « mutilations génitales » en raison de son caractère plus englobant. Il ne s'agit pas ici d'une problématique médicale, mais bien d'une question sociétale qui interroge directement la place des femmes dans la société et leur capacité à disposer de leur corps et à vivre leur sexualité. Aucune tradition culturelle ou religieuse ne saurait justifier ces pratiques profondément ancrées dans la conviction de l'infériorité de la femme et de la fille. Aucun texte religieux ne requiert de telles tortures. C'est une coutume sociétale, parce qu'aucun mari ne voudra d'une épouse non excisée.

pour la première fois dans un manuel scolaire en 2017 ! Nous avons pu mesurer l'ampleur des conséquences effroyables tant physiques que psychiques pour ces femmes, qui sont parfois aggravées par l'infibulation : complications obstétricales, rapports sexuels douloureux, incontinence, douleurs persistantes. Le constat est sans appel : l'excision est bien une torture exercée à l'encontre à l'encontre des femmes et, je le répète, visant à nier l'existence même de leur corps, de leur sexualité et de leur être tout entier. L'une des victimes nous disait : « C'est être vivante et morte à la fois. Nous avons été frappées par le caractère évolutif de ces pratiques. Ces actes de torture sont perpétrés, dans certains pays, par des professionnels médicaux,

et les filles plus âgées sont également concernés aujourd'hui. En France, on vous l'a dit, c'est pendant les congés scolaires, à l'occasion d'un séjour dans leur famille qu'elles risquent d'être excisées, parfois malgré l'avis de leurs parents, parce que c'est la grand-mère

aussi les communautés, les organisations et associations de terrain, les services sociaux et la police, dont les moyens doivent absolument être renforcés. L'engagement résolu des hommes représente également un levier fondamental pour faire évoluer ces pratiques qui ne constituent pas qu'une affaire de femmes, mes chers collègues masculins, mais répondent bien à un ordre établi Ce combat, loin d'être achevé, ne peut être que collectif ! La France a pris conscience de la gravité de l'excision dans les années 1980, notamment lors de la médiatisation de certains procès qui ont fait date. Elle a opposé une réponse pénale forte à ces pratiques, et la loi de 2013 a renforcé la protection des mineurs et les sanctions encourues par les personnes incitant aux mutilations. L'auteur et le responsable de l'enfant mutilé peuvent être poursuivis pour ce type de violences et encourent dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. La France a ratifié en 2014 la convention d'Istanbul du Conseil de l'Europe, laquelle, dans ses articles 37, 38 et 39, exhorte les États parties à éradiquer cette violence. Cette convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique est un instrument juridique exceptionnel qui couvre tout le prisme des violences faites aux femmes et formule de manière pionnière un article très clair pour engager les États à interdire en tant que telles les mutilations sexuelles féminines et pour en faire des infractions pénales. Cependant, la répression ne suffira pas à endiguer cette pratique. Il s'agit aussi de mener des actions d'information et de sensibilisation auprès de chaque professionnel concerné, de chaque communauté, pour faire évoluer les mentalités. Les autorités ont renforcé leur partenariat avec les associations qui offrent aux victimes un soutien matériel et psychologique et qui les aident dans leur parcours d'insertion sociale et professionnelle. Je tiens encore une fois à saluer le travail remarquable qu'elles accomplissent ! La communauté internationale s'en est pleinement saisie à travers un arsenal juridique qui n'a cessé de s'enrichir et nous ne pouvons que nous en féliciter, tant il transcende les frontières et appelle à un engagement collectif et résolu. L'ONU, l'OMS, l'Unicef, sans oublier le travail du comité du prix Nobel de la paix, effectuent chaque jour un travail remarquable pour prendre en charge les victimes et faire évoluer les mentalités et les pratiques par l'éducation. Dès 2001, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, dont je suis membre, a condamné l'excision dans l'une de ses résolutions. En 2013, ma collègue Marlene Rupprecht a réalisé un rapport consacré au droit à l'intégrité physique des enfants. En octobre 2016 est adoptée une résolution sur les mutilations génitales, à la suite du rapport de mes collègues Fresko-Rolfo et Maury Pasquier. Cette dernière est aujourd'hui la présidente de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Ainsi, les efforts conjugués des parlements nationaux et des instances internationales permettent d'enrichir nos réflexions et contribuent à rendre plus visibles ces actes de torture à travers le monde. Malgré une prise de conscience croissante, ces mutilations perdurent et demeurent ancrées dans les cultures et traditions des communautés qui les pratiquent. L'échéance de 2030 fixée par l'ONU pour les éradiquer nous apparaît aujourd'hui bien proche, et il s'agit donc de mener une lutte commune et globale, tant sur le plan législatif qu'éducatif, judiciaire et politique.

la première fois, la participation forte du Sénat à ce combat et à rendre hommage aux professionnels et bénévoles qui, partout dans le monde, oeuvrent au quotidien pour faire avancer les droits des filles, leur accès à l'instruction et partant, la lutte contre les mariages forcés et l'excision. Mes chers collègues, cette cause internationale appelle votre pleine et entière adhésion.

bien qu'ils soient inscrits dans nos lois et dans nombre de conventions internationales, les droits des femmes à disposer de leur corps et à s'émanciper du patriarcat ne sont pas acquis. Ce triste constat ressort régulièrement des travaux de notre délégation. La convention de l'ONU pour l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard des femmes, ratifiée par la France en 1979, statue dans son article 16 que les fiançailles et les mariages d'enfants n'ont pas d'effets juridiques. La convention du Conseil de l'Europe, dite convention d'Istanbul, sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique a été ratifiée en 2011 par trente-trois États dont la France. Son article 38 porte sur les mutilations génitales féminines et l'article 37 oblige les États à voter des lois pour ériger en infraction pénale le fait de forcer un adulte ou un enfant à contracter un mariage ou de le conduire dans un autre État que celui où il réside dans l'intention de le faire. Enfin, en juin 2018, à Charlevoix au Québec, les États du G7, dont la France, se sont engagés à mettre fin à la violence fondée sur le sexe et le genre, ainsi qu'aux abus et au harcèlement dans l'univers numérique, dans l'objectif de promouvoir l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes et de garantir le respect des droits de la personne. Pour atteindre ce but, ils recommandent notamment l'accès de toutes à une scolarité d'une durée minimale de douze années ou encore la levée des obstacles à une éducation de qualité pour les filles. Ils affirment qu'éradiquer la violence faite aux filles est une responsabilité commune, pour laquelle tous ont un rôle à jouer, y compris les hommes et les garçons. garçons. Pour le sommet du G7 prévu à Biarritz en août prochain, la France a défini cinq objectifs pour lutter contre les inégalités, dont l'accès à l'éducation et à la santé. Les auteurs de la proposition de résolution dont nous débattons ont voulu s'inscrire dans cette dynamique. Notre pays a la responsabilité de lutter contre les mariages forcés, les grossesses précoces, les mutilations sexuelles féminines, et c'est à l'unanimité, je tiens à le souligner, que les membres du groupe du RDSE ont décidé de cosigner ce texte. Sans volonté d'ingérence dans les affaires publiques hors de nos frontières, nous rappelons ainsi l'ensemble des mesures à mettre en oeuvre en France pour agir efficacement contre ce fléau, libérer la parole des victimes et les protéger. Le premier pas à franchir était de nommer ces actes pour être mieux en mesure de les combattre. Depuis vingt ans déjà, les victimes parlent, tout comme les acteurs sociaux et les médecins. La prise de conscience est mondiale grâce à des pionniers comme Waris Dirie, devenue l'icône mondiale de la lutte contre l'excision et les mariages forcés, ou encore Denis Mukwege, prix Nobel 2018, Ghada Hatem, gynécologue-obstétricienne ayant installé la Maison des femmes et la chanteuse malienne Inna Modja, elle-même excisée à l'insu de ses parents. Autant de lanceurs d'alertes qui consacrent leur vie à la prévention et au soutien des victimes. Le 11 mars dernier, par exemple, pour la première fois au Royaume-Uni, une femme a été condamnée pour avoir excisé sa fille alors qu'une loi l'interdit depuis 1985. Aujourd'hui, la honte et la peur doivent changer de camp. Lever le voile sur le tabou des mariages forcés, des grossesses précoces et des mutilations sexuelles féminines, c'est aussi reconnaître les souffrances physiques et psychologiques qui laissent dans les chairs des séquelles à vie, parfois innommables pour les victimes elles-mêmes. Malheureusement, ce n'est pas seulement en temps de guerre ou en zone de conflits que les violences sexuelles envers les femmes et les filles sont perpétrées. C'est aussi le quotidien des 200 millions de femmes excisées à travers le monde, dont 60 000 en France. Et ces statistiques sont certainement sous-évaluées Combien dénombrerons-nous encore de victimes de cette tradition, dont le geste technique est perpétré par autant de femmes se conformant au du patriarcat ? Dans notre pays, l'arsenal législatif est solide. L'auteur d'une mutilation s'expose à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. Mais la loi ne suffit pas à changer les mentalités et les injonctions sociales. Après des procès médiatisés dans les années 1980 à 2005, aucune condamnation n'a plus été prononcée depuis 2012. Est-ce à dire qu'il n'y a plus de cas en France ? Ce n'est pas le constat des réseaux associatifs et des professions médicales. Au-delà des chiffres, je veux souligner le rôle de prévention que doivent jouer les équipes éducatives dans les établissements scolaires français, du primaire au lycée. L'éducation à la connaissance de son corps, à la vie sexuelle et reproductive, à la liberté de choisir et au droit universel de disposer de son corps est centrale. Un effort de formation doit être fait à destination des personnels éducatifs et médico-sociaux. Une politique publique de soutien financier aux associations de terrain doit être réaffirmée pour inciter inlassablement les populations à refuser des traditions contraires à la loi, aux droits humains universels et aux conventions internationales, tout simplement parce qu'elles sont criminelles. C'est ainsi, grâce à l'éducation dès le plus jeune âge, que nous gagnerons cette bataille dans les mentalités. De même, il est de la responsabilité du législateur d'être vigilant à chaque instant dans ce domaine. Le Sénat a lancé récemment une mission commune d'information pour lutter contre la pédocriminalité. À ce titre, j'estime que lutter contre les mariages forcés, les grossesses précoces et les mutilations sexuelles féminines, notamment pour ce qui concerne les violences sexuelles perpétrées envers les fillettes et les jeunes femmes mineures encore sous l'emprise du cercle familial, aussi lutter, pour une part, contre la pédocriminalité. N'ayons pas peur des mots, appelons un chat un chat : ces atteintes à leur intégrité physique les privent du plaisir sexuel, bien sûr, mais engendrent aussi des risques pour leur santé, qu'il s'agisse

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la résolution que nous examinons aujourd'hui s'inscrit dans la tradition du Sénat, qui, dès 2006, était à l'initiative d'une loi interdisant le mariage pour les moins de 18 ans.

Aujourd'hui encore, des mutilations sexuelles féminines menacent les jeunes filles en Afrique, mais aussi en Asie du Sud-Est ou, plus près de nous, sur le sol français. Aujourd'hui encore, à La Réunion, mais ailleurs également, les grossesses précoces restent une menace à l'épanouissement plein d'une vie de femme. Cette résolution, vous l'aurez compris, dépasse le cadre de notre assemblée et nous rappelle que la France a pour devoir d'éclairer les consciences. « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres

Car, même si les modalités sont différentes, le mariage des enfants, les grossesses précoces et les mutilations sexuelles féminines relèvent d'une même logique et ont,, les mêmes conséquences.

L'objectif est toujours le même, quelle que soit la forme de violence pratiquée : nier le corps de la femme, étouffer sa parole et lui refuser l'envol de l'esprit en lui refusant l'éducation. C'est bien là une forme de servilité. Malala, cette jeune Pakistanaise, nous a rappelé voilà quelques années que certains sont prêts à tuer pour laisser les jeunes femmes dans l'ignorance. Et Nassimah, pour avoir été mariée à 17 ans au sein de la République française, peut vous dire que certains parents pensent bien faire quand ils agissent en perpétuant leurs propres traditions et croyances ... L'école, l'éducation, est la seule voie pour s'extraire des chemins tout tracés par les familles, les traditions ou les religions pour les adolescentes d'hier et d'aujourd'hui. Quels que soient les pays, les conséquences de ces pratiques sont toujours les mêmes. Elles sont psychologiques, sanitaires, avec une surmortalité des femmes, notamment lors des accouchements. Elles sont sociales, avec des sociétés rigidifiées, sans évolution possible. Elles sont économiques, enfin, puisque ces pays, en se privant des femmes, se privent d'une partie de leur richesse et de leur potentialité de développement.

comme cette plateforme nationale des religieux mise en place en Guinée sous la houlette de la ministre de l'action sociale et de la promotion féminine, agir en soutenant des projets de coopération avec les pays les moins avancés, car le mariage des enfants reste étroitement associé à la pauvreté. Dans beaucoup de pays, une fille est souvent considérée seulement comme une bouche à nourrir. La grande dame que fut Simone Veil aurait été honorée de voir, le 8 mars dernier, que le premier prix qui porte son nom a été remis par le Président de la République à Aïssa Doumara, une activiste camerounaise qui lutte contre les mariages forcés et les violences faites aux femmes.

pouvoir tout dire du monde, nous ne dénonçons pas ces agissements condamnables, alors même que ces combats font partie des objectifs du millénaire pour le développement. Je me rappelle par exemple des confidences de ces adolescentes aux Comores, me demandant que cessent les abus de certains, des des maîtres d'école coranique agissant en toute impunité. Je porte leur parole sur mes épaules. Je pense aussi à l'Éthiopie, où 75 % des petites filles sont encore excisées. Chers collègues, cette résolution nous rappelle à ce devoir moral de dénonciation

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, « tant que les femmes et les filles, qui forment la moitié de la population de la planète, ne vivront pas à l'abri de la peur, de la violence et de l'insécurité quotidiennes, il nous sera impossible de prétendre vivre dans un monde juste et égal ». Tout est dit dans cette phrase prononcée par Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. Mais il y Mais il y a les paroles, et les actes. Les paroles, ce sont les dénonciations, c'est ce que nous faisons aujourd'hui avec cette résolution, que le groupe Les Indépendants soutient, dénoncer que plus d'une femme ou une fille sur trois est victime de violence au cours de sa vie, que 750 millions de femmes ont été mariées avant l'âge de 18 ans et que plus de 250 millions d'entre elles ont subi des mutilations génitales. Aujourd'hui, la violence à l'égard des femmes et des filles constitue l'une des violations des droits de l'homme les plus répandues, les plus persistantes et les plus dévastatrices dans le monde. Et malheureusement, la lutte contre les mutilations n'est pas sur le point de s'achever : les chiffres sont en hausse et les prévisions sont mauvaises. Pourtant, rien ne saurait justifier cette pratique barbare, même si certains s'y risquent et avancent des motifs d'hygiène, évidemment absurdes quand on sait les conditions sanitaires dans lesquelles cette mutilation est effectuée. Et je ne parle pas des conséquences médicales, qui vont de l'hémorragie au risque accru de décès lors de l'accouchement, en passant par de fréquentes et insupportables douleurs. Dénoncer, nous le faisons, encore et encore, et nous devons continuer. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut agir Agir, c'est ce qu'a fait Waris Dirie, jeune somalienne qui a pu échapper à l'âge de 13 ans au mariage arrangé par son père. Devenue mannequin international, elle a été nommée ambassadrice de bonne volonté pour l'ONU après avoir raconté dans les médias le drame de son excision à 5 ans. le destin hors du commun d'une femme qui a profité de sa célébrité pour défendre les droits des femmes., un film poignant réalisé d'après son oeuvre originale, a été programmé par Arte la semaine dernière à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Agir, c'est le combat mené par Aïssa Doumara Ngatansou depuis plus de vingt ans au sein de l'Association de lutte contre les violences faites aux femmes, l'ALVF, après avoir dit non à 15 ans au mariage forcé au Cameroun. Elle vient de recevoir le premier prix Simone-Veil de la République française, favorisant des actions en faveur du droit des femmes. Mais nous savons que des centaines de milliers de Waris et d'Aïssa bravent chaque jour les préjugés sexistes et certaines traditions bien ancrées pour prendre le chemin de la liberté, de la connaissance et d'un avenir meilleur, au péril de leur vie. Agir, c'est le combat mené par Denis Mukwege, le gynécologue congolais surnommé « l'homme qui répare les femmes », et qui a remporté le prix Nobel de la paix. Agir, c'est l'initiative Spotlight, partenariat entre l'Europe et l'ONU, qui déploiera des investissements ciblés à grande échelle en Asie, en Afrique, en Amérique latine, dans le Pacifique et dans les Caraïbes, avec pour objectif d'obtenir des améliorations importantes dans la vie des femmes et des filles. Agir, c'est une décision prise la semaine dernière par le Royaume-Uni, qui vient de condamner à onze ans de prison une femme ougandaise pour l'excision de sa fille de 3 ans. Au moment des faits, elle avait invoqué une simple chute dans la cuisine pour expliquer la blessure de son enfant. Mes chers collègues, ces pratiques que nous dénonçons aujourd'hui nous concernent aussi, nous Français. D'abord parce que 60 000 femmes et filles mutilées à l'étranger vivent en France. Notre premier devoir est de convaincre nos concitoyens que ces mutilations sont inacceptables. Il nous faut ensuite les combattre afin que plus aucune de nos filles ne risque de les subir. Je veux saluer l'engagement de Marlène Schiappa pour la lutte qu'elle mène contre le mariage forcé et l'excision. En effet, ne l'oublions pas, la loi française interdit l'excision et protège toutes les filles qui vivent en France, quelle que soit leur nationalité et quel que soit le territoire où elle est pratiquée. La loi condamne également le fait de contraindre une personne à se rendre à l'étranger pour l'y marier de force, notamment en lui cachant le vrai motif de son voyage. Au-delà du combat pour la justice et contre les discriminations, la scolarisation des filles est également, à mon sens, une réponse. La privation d'instruction enferme les filles, puis les adolescentes et les femmes qu'elles seront, dans une extrême vulnérabilité face à la maladie, au sida, aux violences sexuelles, aux mariages forcés, aux grossesses précoces et à la pauvreté. Aujourd'hui encore, 64 millions de filles âgées de 6 à 14 ans n'ont pas accès à l'éducation. Et comme l'a dit Kofi Annan, « il n'existe aucun instrument de développement plus efficace que l'éducation des filles Une fille éduquée peut plus facilement faire entendre sa voix, a plus de facilités à accéder et à suivre les recommandations et conseils de prévention et de soins pour elle-même et ses enfants, comprend l'intérêt de donner à ses enfants une éducation de qualité, ose résister à un projet de mariage précoce et connaît l'existence de moyens de contraception. Alors, parce que ces actes, dirigés contre les femmes, portent atteinte à la dignité humaine, la France doit se montrer à la hauteur de son histoire et se doit de faire entendre sa voix. Un discours antiféministe jusque-là en sommeil refait surface en Europe. L'égalité entre les femmes et les hommes est remise en cause en Hongrie, le droit à l'avortement est menacé en Pologne. Il nous faut garder une vigilance de tous les instants face à ces menaces, comme il nous faut faire de ce combat contre les violences faites aux femmes le combat du XXI siècle. C'est l'honneur de la France et des Français que de mener ce combat aussi longtemps qu'il le faudra. Pour conclure, je félicite et remercie la délégation aux droits des femmes, sa présidente Annick Billon

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, au lendemain de la Journée internationale des droits des femmes et de la remise du prix Simone-Veil à la Camerounaise Aïssa Doumara, qui, à travers son association, vient en aide aux victimes de viols et de mariages forcés dans son pays, la délégation aux droits des femmes nous invite à débattre de la proposition de résolution pour soutenir la lutte contre le mariage des enfants, les grossesses précoces et les mutilations sexuelles féminines. Cette proposition de résolution s'inscrit dans la continuité des travaux de la délégation aux droits des femmes. Les mutilations sexuelles, les mariages forcés et les grossesses précoces touchent aux droits fondamentaux des femmes et des enfants. Aucune tradition ne saurait justifier des pratiques barbares qui bafouent les droits des enfants et des femmes. Les statistiques terribles ont été rappelées, mais elles méritent d'être martelées : toutes les sept secondes dans le monde, une jeune fille de moins de 15 ans est mariée contre son gré une fille sur cinq met au monde son premier enfant avant l'âge de 18 ans ; plus de 70 000 décès sont causés chaque année par les grossesses et les accouchements précoces. Le mariage forcé n'est pas une violence isolée. Il faut rappeler que le mariage forcé des jeunes filles revient à un viol conjugal permanent, dont il faut aussi souligner les dimensions pédophiles aggravantes. Dans le cadre du mariage forcé, les filles sont considérées comme monnaie d'échange, soumises au bon vouloir des hommes. En privant les filles de scolarisation, elles sont empêchées de s'émanciper un jour de la tutelle des hommes. La scolarisation et l'éducation des filles comme des garçons restent le meilleur moyen de retarder et de prévenir le mariage des enfants. Il est donc indispensable d'investir massivement dans une éducation de qualité pour les filles, notamment pour les plus défavorisées. Le mariage précoce et forcé persiste, voire se développe dans les régions en crise où la détresse économique et sociale a des conséquences dramatiques sur la situation des enfants. Il existe un entre mariage des enfants et mutilations sexuelles féminines : selon de nombreux témoignages, il est fréquent qu'une très jeune fille subisse une excision pour être ensuite mariée de force. Les statistiques mondiales des mutilations sexuelles féminines sont tout aussi dramatiques que celles des mariages précoces. Toutes les quinze secondes dans le monde, une fillette ou une femme est excisée. Le nombre de victimes s'élève actuellement à 200 millions, dont 44 millions ont moins de 15 ans. Il s'agit donc véritablement d'une violence faite aux femmes et aux enfants. Face à ces terribles constats, la proposition de résolution souligne que l'inscription à l'état civil d'un enfant est un droit fondamental qui conditionne la réalisation d'autres droits. À défaut, une personne qui n'est pas déclarée à l'état civil peut être exposée à toutes sortes de trafic. La proposition de résolution rappelle que, en 2006, sur l'initiative du Sénat, le mariage au-dessous de l'âge de 18 ans a été interdit, pour les filles comme pour les garçons- cette règle peut avoir valeur d'exemple pour tous les pays engagés dans la lutte contre les mariages précoces. Elle manifeste son soutien aux acteurs de la lutte contre le mariage des enfants et les mutilations sexuelles féminines et souhaite que les moyens qui leur sont attribués soient à la hauteur des besoins. Monsieur le secrétaire d'État, les subventions attribuées par la France aux associations investies dans la lutte contre le mariage forcé et les mutilations sexuelles féminines devraient faire l'objet d'un effort spécifique et être sanctuarisées dans un cadre pluriannuel. Les personnels scolaires se trouvent en première ligne pour contribuer au repérage et à l'orientation des victimes potentielles. La proposition de résolution appelle à sensibiliser les personnels de l'éducation nationale, y compris les infirmières, les psychologues et les médecins scolaires aux risques encourus par les jeunes filles qui, à l'occasion d'un séjour dans le pays d'origine de leur famille, pourraient être excisées et mariées de force. Les moyens de la médecine scolaire doivent donc être renforcés pour mettre en oeuvre un meilleur repérage des victimes et la protection des petites filles et des adolescentes contre l'excision et le mariage précoce. La proposition de résolution appelle de ses voeux que la diplomatie française continue à mettre l'accent sur le caractère crucial de l'accès à l'éducation pour toutes les filles, et qu'elle soit particulièrement attentive au sort des fillettes, des adolescentes et des femmes dans les régions en crise. Monsieur le secrétaire d'État, nous comptons sur un engagement fort de notre pays pour protéger les enfants et les jeunes filles dans ces régions. Enfin, je tiens à remercier la présidente de la délégation aux droits des femmes de nous donner l'occasion de débattre de la lutte contre les mariages forcés, les mariages des enfants et les grossesses précoces. Je profite de cette occasion pour saluer également le travail remarquable de mes collègues Marta de Cidrac et Maryvonne Blondin.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, chaque année, 12 millions de filles sont mariées avant l'âge de 18 ans, parfois même avant 11 ans. Le partenaire leur est imposé, et il est souvent beaucoup plus âgé qu'elles. Après le mariage vient la grossesse, souvent forcée elle aussi. La femme doit faire autant d'enfants que le souhaite son mari, et ce malgré les risques dus à son jeune âge. En effet, les grossesses précoces causent 70 000 morts chaque année. Les complications liées à la grossesse et à l'accouchement sont la deuxième cause de décès dans le monde pour les filles de 15 ans à 19 ans. Le mariage des enfants et les mutilations sexuelles sont liés. Il est fréquent que les jeunes filles subissent une excision pour être ensuite mariées. Et les chiffres sont tout aussi effroyables : toutes les quinze secondes dans le monde, une fillette ou une femme est excisée. Le nombre de victimes s'élève aujourd'hui à 200 millions, dont le quart a moins de 15 ans. Les conséquences de l'excision sur la santé physique et psychologique des femmes sont graves. Lorsque ces mutilations sexuelles sont pratiquées sur de jeunes enfants, avant l'âge de 3 ans, c'est 10 % à 15 % de mortalité immédiate. C'est le fait de croyances religieuses, de traditions et de conceptions des rapports entre les sexes considérant les femmes non seulement comme des objets, mais aussi comme propriétés des hommes. En France, l'excision est fermement condamnée. Mais nous savons que des adolescentes vivant sur notre territoire en sont menacées lors de séjours dans le pays d'origine de leur famille. Outre la défense des cultures et des traditions, un illusoire prétexte d'hygiène est parfois invoqué. Il est inacceptable de constater un tel dévoiement de la profession au profit de pratiques religieuses et traditionnelles. Aussi est-il impératif de lutter contre tout type de croyance cherchant à justifier ces mutilations. Mariages forcés, grossesses précoces, mutilations sexuelles sont autant de violations des droits fondamentaux. Dans certains pays, ces crimes sont perpétrés dans des situations de conflit armé ou d'après-conflit et, dans la plupart des cas, les individus qui les ont commis ne seront pas jugés. Cette impunité ne saurait être tolérée. Nous devons condamner ces violences par tout moyen dont nous disposons. Dans la lutte pour l'égale dignité des femmes et des hommes, nous sommes tous concernés, et l'implication des hommes est tout aussi décisive. Il est de notre devoir de renforcer la protection des mineurs. Il y va de la liberté pour chacun de disposer de son corps et de sa propre vie il y va du droit à l'enfance et du droit à l'éducation pour toutes et tous. Cette proposition de résolution rend également hommage à toutes celles et tous ceux qui s'engagent dans le combat contre ces sévices. Je pense, entre autres, à Denis Mukwege, ce gynécologue congolais surnommé « l'homme qui répare les femmes » et à Aïssa Doumara Ngatansou, militante camerounaise à qui le Président de la République a remis le premier prix Simone-Veil le 8 mars dernier, à des ONG ou encore à des organisations internationales telles que l'Unicef. Prenons exemple sur ces personnes pour lutter contre les exactions et promouvoir l'éducation des jeunes filles, qui permet de lutter contre la mortalité maternelle et infantile. Par cette proposition de résolution, le Sénat rejoint la résolution du Parlement européen du 23 mars 2009 sur la lutte contre les mutilations génitales féminines. Je m'en réjouis. La chambre haute, trop souvent considérée comme conservatrice, et sa délégation aux droits des femmes, composée de sénateurs de tous bords, démontrent ainsi un engagement commun pour défendre les droits fondamentaux des femmes. Pour ces raisons, le groupe La République En Marche votera en faveur de cette proposition de résolution pour lutter contre le mariage des enfants, les grossesses précoces et les mutilations sexuelles féminines. OEuvrons à l'égale dignité des femmes et des hommes partout dans le monde, et pour que la France soit considérée comme le pays des droits des hommes et des femmes. Enfin, je tiens à remercier les auteures de la proposition de résolution.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, à mon tour, je voudrais remercier la présidente de la délégation aux droits des femmes, Annick Billon, et nos deux corapporteures, Marta de Cidrac et Maryvonne Blondin, de nous avoir permis de mener un travail très approfondi sur ces enjeux de violation des droits des filles et des femmes. À la suite de ce travail, il me paraît effectivement essentiel que la Haute Assemblée prenne position contre les mutilations sexuelles en approuvant cette proposition de résolution, que j'ai cosignée avec l'ensemble de mes collègues du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

la répétition est pédagogique, paraît-il. Ainsi, 160 millions de femmes sont mutilées à travers le monde, dans 85 pays, et 3 millions de fillettes encourent un risque chaque année. En France, un peu plus de 60 000 femmes sont concernées. 12 millions de filles sont mariées chaque année dans le monde avant l'âge de 18 ans, qu'une fille sur cinq donne naissance à son premier enfant avant 18 ans et que 70 000 décès sont causés chaque année par les grossesses et accouchements précoces. Ces chiffres sont terribles et démontrent, s'il en était besoin, le des violences dont sont victimes ces fillettes et ces jeunes filles. La cause principale de ces violences est la domination masculine, le système patriarcal qui sévit partout dans le monde. Notre rôle de législateur est de dénoncer et de lutter contre ce système de violences de genre qui infériorise les femmes et va jusqu'au plus profond de leur chair, s'immisçant dans leur intimité en leur interdisant tout désir et tout plaisir sexuels. Ces mutilations sexuelles féminines sont l'expression de l'appropriation du corps des femmes par les hommes. J'ai encore en mémoire le déplacement que

publié par l'une d'entre elles, Mme Diaryatou Bah ? Comment oublier le cri de douleur, au sens propre, qu'elles ont relayé et qui résonne en elles comme en nous ? Je tiens donc à saluer l'engagement des associations qui oeuvrent au quotidien- je pense notamment au GAMS et à Excision, parlons-en

fassent l'objet, comme celles de toutes les associations engagées contre les violences faites aux femmes, d'un effort spécifique, dans un cadre pluriannuel Outre cet appui aux associations qui se battent au quotidien auprès des femmes mutilées, il est nécessaire de mener et de développer des campagnes de communication, singulièrement à destination des jeunes qui doivent être informés et sensibilisés. Il nous faut également être très attentifs aux moyens accordés à la Cimade et aux conditions de travail des agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de ceux de l'aide sociale à l'enfance. Toutes ces structures sont indispensables pour repérer les violences et accompagner les jeunes filles au plus tôt. Évidemment, le corollaire, c'est la nécessité de former tous les professionnels qui sont en lien avec les enfants et les adolescents : médecins scolaires- enfin, ce qu'il en reste ! -, infirmières, assistantes sociales ... C'est notamment pourquoi je regrette,

Sur le plan international à présent- notre proposition de résolution l'évoque -, il est impératif que de nombreux pays s'engagent à signer la convention d'Istanbul, ratifiée par la France en 2014 et qui comprend notamment l'article suivant : « Les parties veillent à ce que la culture, la coutume, coutume, la religion, la tradition ou le prétendu " honneur " ne soient pas considérés comme justifiant des actes de violence couverts par le champ d'application de la présente convention. » Pourquoi ne pas profiter de la présidence française du G7, à partir d'août 2019, pour faire avancer la question de l'accès à l'éducation pour toutes les filles, pour interdire dans tous les pays le mariage pour les filles comme pour les garçons au-dessous de 18 ans et pour engager les États à interdire, en tant que telles, les mutilations sexuelles féminines et en faire des infractions pénales Car toutes les personnes que nous avons rencontrées, notamment lors de l'audition de l'Unicef, nous ont bien confirmé que les conséquences de ces violences sont multiples : les petites filles ne vont pas ou plus à l'école, elles souffrent terriblement et vivent par la suite dans une dépendance et une précarité économique évidentes, toutes connaissent des problèmes de santé

De même, pouvez-vous nous en dire davantage sur l'engagement du Président de la République de créer dix lieux de soins innovants dans ce domaine ? Je terminerai mon propos en citant le Dr Mukwege, prix Nobel de la paix, que j'ai eu l'honneur de rencontrer récemment : « Je Je voudrais vous dire qu'à travers ce prix le monde vous écoute et refuse l'indifférence. C'est vous, les femmes, qui portez l'humanité

le 11 octobre 2018, le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, Antonio Guterres, disait : « En cette Journée internationale de la fille, engageons-nous de nouveau à aider chaque fille à développer ses compétences, à entrer dans le monde du travail sur un pied d'égalité et à exploiter tout son potentiel. » Une fois encore, il rappelait que le chemin à parcourir reste long en matière d'éducation ou de santé, mais aussi dans les mentalités, y compris Ces engagements ne sont pas sans rappeler le 6 février, Journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines, qui a été instituée par une résolution de l'Organisation des Nations unies en 2012. de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, à laquelle j'appartiens depuis le renouvellement du Sénat de septembre 2017, nous avons voulu mettre l'accent sur les fléaux que sont le mariage des enfants, les grossesses précoces et les mutilations

une fillette ou une femme est excisée ; une fille sur cinq donne naissance à son premier enfant avant l'âge de 18 ans ; 70 000 décès dans le monde sont causés chaque année par des grossesses précoces.

par des traditions culturelles ou religieuses. Ces pratiques illustrent, mes chers collègues, la place que l'on donne à la femme, à l'enfant et tout simplement à l'humain dans la société. Je tiens à remercier

La qualité de ces travaux et les différentes auditions et tables rondes qui se sont tenues nous permettent, aujourd'hui, de réaffirmer notre mobilisation face aux fléaux que vivent les femmes et les jeunes filles.

L'ensemble de ces dispositifs a un coût, et nous ne pouvons mener ces combats sans moyens financiers suffisants. C'est pourquoi nous recommandons que des subventions soient attribuées par la France aux différentes associations investies dans la lutte contre le mariage forcé

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je tiens d'abord à féliciter Annick Billon, présidente de la délégation aux droits des femmes du Sénat, Marta de Cidrac et Maryvonne Blondin d'avoir été à l'initiative de cette proposition de résolution, que j'ai bien évidemment cosignée. Je tiens également à féliciter les associations qui luttent contre le mariage des enfants et les mutilations sexuelles féminines. Les grandes vacances en famille dans les pays d'origine des parents devraient être source de bonheur, de joie et d'insouciance pour les petites filles et les adolescentes. Las, pour certaines, elles deviennent un cauchemar. On ne peut ni tolérer l'intolérable ni accepter l'inacceptable. Traiter les femmes comme des humains de seconde zone est une tradition inacceptable. Les pratiques de l'excision et du mariage forcé sont inexcusables au XXI siècle et n'ont aucune place dans une société civilisée. Si les mariages forcés entre adultes sont une réalité, nombre d'entre eux sont imposés à de jeunes filles, voire à de petites filles. Les chiffres mentionnés dans la proposition de résolution sont édifiants. Derrière ces tristes chiffres se cachent autant de vies brisées, de talents et potentiels gaspillés et de risques graves pour la santé, sur le plan tant psychique que physique. Un mariage précoce entraîne le plus souvent un abandon de la scolarité, un passage trop rapide à la vie d'adulte, une enfance volée, un esclavage domestique, des relations sexuelles subies et des grossesses non désirées et dangereuses pour la santé. Nous abordons le sujet de manière abstraite, habitués- malheureusement presque anesthésiés -par la vie et nos activités parlementaires à traiter de sujets graves. Mais projetez-vous dans votre passé, mes chers collègues, et imaginez que vous ayez été mariés de force à l'âge de 15 ans Dans des camps de réfugiés, c'est même à 11 ans que certaines petites filles sont mariées afin d'obtenir des rations alimentaires et une protection. On observe, hélas ! une corrélation logique entre multiplication des conflits et des catastrophes naturelles, d'une part, et augmentation des mariages forcés, d'autre part. Ces explications de détresse et d'urgence vitale ne sont pas les seules raisons. Il faut aussi changer les mentalités : dans certains pays du monde, nombreux sont les parents qui, n'ayant pas les moyens d'offrir une éducation à leurs enfants, estiment que la solution est de les marier.

car elle permet d'agir. En effet, il arrive que, lorsque des témoins osent parler, un mariage soit annulé et que la jeune fille puisse être rescolarisée. Si parfois les campagnes de prévention sont bien accueillies, il n'est pas rare qu'elles se heurtent à la résistance des différents corps sociaux des communautés, où la pratique est bien ancrée, ainsi qu'à celle des parents. En ce qui concerne les mutilations sexuelles féminines défendues par les femmes elles-mêmes, elles sont vues comme un acte d'honneur dans des sociétés qui considèrent que le corps de la femme est la propriété des hommes de la famille. Le rapport de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, dont je suis membre, fait observer que « les normes sociales jouent un rôle clé dans la persistance de ces pratiques : elles sont la marque d'une culture et d'une tradition, dont le non-respect entraîne nécessairement le rejet social et la marginalisation Comme cela est souligné dans le rapport d'information fait au nom de la délégation aux droits des femmes du Sénat par nos collègues Maryvonne Blondin et Marta de Cidrac, dont je salue l'excellent travail, le Dr Ghada Hatem explique que cette idée de rite initiatique est tellement ancrée dans la tête des petites filles qu'elles pensent être impures si elles n'en passent pas par là. Le plus dramatique est certainement le fait que le corps médical se prête parfois à ces pratiques, sous le prétexte d'offrir des conditions d'hygiène optimales. Je me réjouis que le Sénat prenne part à la mobilisation, dans laquelle s'est déjà inscrit le Conseil de l'Europe avec les résolutions 2233, adoptée en 2018 sur les mariages forcés en Europe, et 2135, adoptée en 2016 sur les mutilations génitales féminines en Europe.

à l'intégrité physique. Il avait aussi appelé les États membres à intégrer de manière systématique les mutilations génitales féminines dans les procédures et politiques nationales de lutte contre les violences, ainsi qu'à mener des campagnes de sensibilisation contre ces violences, notamment en fournissant des informations dans les langues les plus parlées par les communautés pratiquant ces mutilations. Ayez conscience, chers collèges, que nous serons jugés par nos enfants, non seulement sur ce que nous aurons réalisé, mais aussi sur ce que nous n'aurons pas fait ! Il est donc de notre devoir de faire tout notre possible, de mettre toutes nos forces dans cette lutte et de saisir toutes les marges de manoeuvre, aussi faibles soient-elles, pour éviter que perdurent ces pratiques barbares qui ne sont pas dignes de l'être humain. La différence de nos cultures, loin de nous éloigner, nous enrichit dans la limite, néanmoins, du respect et de la dignité qui sont dus à la personne humaine. Je voterai bien entendu cette

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, à Lille-II, il y a quelques années, la faculté de droit avait décidé d'ouvrir un master de droit consacré à la direction des structures dans le champ social. J'en étais le professeur de droit de la famille. Quelques étudiants avaient choisi de s'intéresser, pour leur stage de validation d'études, à la problématique des grossesses précoces dans le Nord, nombreuses selon les statistiques. Les étudiants voulaient rencontrer les jeunes filles concernées afin d'étudier leurs difficultés et voir comment les assistantes sociales pouvaient leur apporter une aide personnalisée et leur donner une chance de sortir de la précarité. À leur grand étonnement, les équipes éducatives les ont dirigés vers les collèges. Eh oui, c'est bien dans des collèges que ces étudiants ont pu rencontrer des filles en situation de grossesse précoce Je me souviendrai toujours de cette anecdote glaçante, et je souhaitais la partager avec le Sénat et avec vous, monsieur le secrétaire d'État. Conseillère générale, je me rendais très souvent dans les foyers de mères enfants du Nord. J'y ai vu des jeunes filles en grande précarité, confrontées au plus grand des défis : être mère. Certaines d'entre elles avaient même deux petits lits dans leur chambre, un à barreaux et un berceau. Beaucoup étaient protégées pour elles-mêmes en tant que mineures en danger et leur propre enfant faisait aussi l'objet d'une protection judiciaire d'assistance éducative.

Ayons une pensée pour toutes les petites Françaises nées ce jour ! Quel sort sera réservé à Marie, à Sarah ou à Inès ? La logique voudrait qu'elles soient égales en tout point à leurs compatriotes masculins, tous les citoyens naissant libres et égaux en droits en France ... Si elles étaient nées ailleurs sur le globe, elles auraient pu subir des mutilations sexuelles moyenâgeuses, telles que l'excision.

plus de 60 000 femmes ayant subi cette pratique vivent en France de nos jours et près de 500 000 dans toute l'Union européenne. Et ces chiffres croissent chaque année ! Comment l'accepter ? Encore en France, près de 70 000 de nos jeunes filles vivraient dans la crainte d'un mariage forcé. La présente proposition de résolution pour soutenir la lutte contre le mariage des enfants, les grossesses précoces et les mutilations sexuelles féminines est donc indéniablement nécessaire. En France, la législation n'a cessé d'évoluer depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale pour parvenir, en principe, à une égalité des droits entre les femmes et les hommes. Je ne

pour changer les mentalités dans l'Hexagone et au-delà. Un flash d'information circule en ce moment sur les écrans de télévision pour dire qu'il n'y a rien de viril à frapper une fille. J'espère que ce message sera entendu et fera évoluer la mentalité des jeunes garçons. J'ai passé ma vie universitaire à me féliciter de voir des jeunes femmes sortir majors de leurs promotions, rafler les premières places dans des concours prestigieux et s'affirmer dans leurs vies professionnelles. Je ne peux m'empêcher, malgré tout, de m'étonner de leur absence dans les plus hautes sphères de notre société. Le temps a fait son oeuvre et les femmes sont de plus en plus nombreuses à décrocher la place qu'elles méritent, mais cette progression est encore trop lente. Profitons de l'occasion de cette proposition de résolution pour réaffirmer nos principes, nos valeurs, notre richesse la plus fondamentale Car c'est une fois que nous aurons combattu et vaincu nos propres démons que nous pourrons faire entendre de manière forte et fière la voix de la France à l'international,

la Commission nationale consultative des droits de l'homme affirmait, en 2013, que « nul droit à la différence, nul respect d'une identité culturelle ne saurait légitimer des atteintes à l'intégrité de la personne,

53 000 femmes mutilées. En 2016, en France toujours, sur 250 683 filles originaires de pays où les mutilations sexuelles féminines sont pratiquées,

Toutes les sept secondes dans le monde, une jeune fille de moins de 15 ans est mariée contre son gré. En ce 14 mars 2019, vous avez été nombreux à le rappeler, 70 000 décès sont dus chaque année à des grossesses et à des accouchements précoces. En 2019, les complications liées à la grossesse et à l'accouchement sont la deuxième cause de décès dans le monde pour les jeunes filles âgées de 15 à 19 ans. Aucune tradition ne saurait être invoquée pour justifier les mutilations sexuelles féminines qui bafouent les droits fondamentaux des femmes et des petites filles et constituent une violence dont sont victimes tant des femmes que des enfants. Aucune tradition ne saurait être invoquée pour justifier le mariage précoce, qui n'est rien d'autre qu'un mariage forcé, car il est inenvisageable qu'une enfant puisse y consentir librement. Eh oui, évidemment, ces sujets ne concernent pas que les femmes

La lutte contre les mutilations sexuelles féminines est au coeur de l'action du Gouvernement, dont celle de la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, que je souhaite évidemment associer à mes propos. Marlène Schiappa, en écho aux

et des associations. La secrétaire d'État Marlène Schiappa a lancé, à la demande du Premier ministre, des travaux en vue d'élaborer un plan national d'action visant à éradiquer les mutilations sexuelles féminines.

Si l'accent est aujourd'hui mis sur les actions de lutte contre les mutilations sexuelles, celles-ci ont, par ricochet, un effet levier pour lutter contre les mariages précoces et forcés, notamment dans le cadre de la sensibilisation, de la formation et du repérage. Vous avez été nombreuses à soulever Lutter contre ces violences, c'est diffuser, dès le plus jeune âge, le principe d'une égalité entre les femmes et les hommes, d'une égalité entre les filles et les garçons à travers une politique de prévention dans les crèches et les écoles, partout où les enfants apprennent, échangent et se construisent. L'éducation L'éducation est un élément clé de la prévention, comme la médecine scolaire, qui, grâce aux ministères de la santé et de l'éducation nationale, permet de prévenir et de repérer ces violences. Le ministère de la santé, que je représente ici, mène, d'ailleurs, au travers de nombreux projets,

une équipe pluridisciplinaire composée de chirurgiens mais aussi de sages-femmes, de psychologues, d'assistantes sociales et d'infirmières, afin de soutenir ces femmes mutilées en prenant en charge leur douleur et en leur proposant un encadrement en sexologie. Prévenir, parler, accompagner

et je m'en réjouis, du conseil consultatif sur l'égalité entre les femmes et les hommes que nous mettrons en place à l'occasion du G7. Enfin, au niveau international, la France, signataire depuis 2011 de la convention d'Istanbul, a lancé une campagne de promotion de cette convention. Cette campagne pour l'universalisation de la convention d'Istanbul, standard de protection des femmes face aux violences sexistes et sexuelles dans l'Union européenne, appelle tous les États à la ratifier. La présidence à la ratifier. La présidence française du G7 a également mis l'égalité entre les femmes et les hommes au coeur de ses priorités en s'appuyant sur deux objectifs, qu'un certain nombre d'entre vous ont rappelés d'abord, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, dont la lutte contre l'excision et le mariage forcé ; ensuite, l'éducation des femmes, dont le coeur d'action est l'accès des filles à l'école. Oui, je veux rappeler devant vous que chaque fille, chaque femme de notre République a le droit de se marier et de vivre sa sexualité comme elle le souhaite ! En France, vivent 53 000 femmes mutilées. Chaque année, 12 millions de filles sont mariées avant l'âge de 18 ans dans le monde. Combien encore de destins gâchés, d'enfances bafouées faudra-t-il pour que cette violence contre nos enfants prenne fin ? Je salue votre mobilisation ici, ainsi que celle de nombreuses associations- Excision, parlons-en !, GAMS, la maison des femmes,

Nous nous devons d'envoyer un message fort à toutes ces victimes et à tous ceux qui s'engagent pour la lutte contre les mariages forcés, les grossesses précoces et les mutilations génitales. Le travail de Marta de Cidrac et de Maryvonne Blondin doit être souligné. Il a largement précédé les annonces de Mme la secrétaire d'État. Souhaitons qu'elle s'inspire du travail de notre délégation et, plus généralement, de celui du Sénat, souvent en avance sur les sujets, l'actualité sénatoriale de cette semaine l'a encore démontré.

notre institution. Le groupe Les Républicains s'associe bien évidemment au vote de cette proposition de résolution et à la mobilisation qui l'accompagne. En effet, il est essentiel de se mobiliser face à ce fléau de l'asservissement de fillettes à des règles ancestrales, toujours dictées par des hommes. Les mariages précoces et forcés, les excisions, qui se pratiquent encore dans une trentaine de pays, ne sont pas tolérables. tolérables. Ni la culture ni la religion ne sauraient justifier la violence faite aux victimes. C'est justement parce que la barbarie est entrée, il y a des siècles, dans les traditions familiales, parce qu'elle se transmet même de mère en fille, que notre société doit la rejeter avec la plus grande fermeté et tout faire pour entraver ces pratiques. Les chiffres qui ont été évoqués- une fillette de moins de 15 ans mariée toutes les sept secondes dans le monde, une fillette excisée toutes les quinze secondes -montrent l'ampleur du désastre et, donc, l'intérêt de toute pierre apportée à l'édifice. Cette proposition de résolution rend hommage aux bénévoles et professionnels qui oeuvrent au quotidien dans le monde entier. Elle dresse un bilan des actions déjà menées aux niveaux international et européen. de résolution n'est pas qu'une déclaration de principes. En mettant en oeuvre plusieurs recommandations du rapport de nos collègues Maryvonne Blondin et Marta de Cidrac, elle appelle le Gouvernement à approfondir son action. L'accueil de populations immigrées implique en effet une vigilance accrue. Ainsi, nous demandons un effort financier renforcé et pluriannuel vers les associations et la sensibilisation de tous les acteurs de la vie quotidienne qui pourraient être amenés à repérer, signaler ou orienter une victime. Comme il a été souligné, l'éducation nationale joue un rôle majeur dans la prévention et le signalement de cas. Il faut donc assurer une meilleure formation des personnels et renforcer les moyens de la médecine scolaire. Monsieur le secrétaire d'État, nous comptons également sur l'influence française et sa présidence à la tête du G7 pour que soit encore amplifiée

Le scrutin est ouvert.

Le Sénat a adopté.